prévoyait des solutions pour régler bien des problèmes dans des territoires subissant depuis trop longtemps des situations de désordre foncier, en premier lieu en Corse. Il existe dans notre pays un désordre de la propriété lié à l’absence de titres opposables, à l’existence de biens non délimités dont on ne connaît pas exactement les droits qu’il s’agisse des droits de chacun des propriétaires présumés ou encore de l’existence de comptes cadastraux appartenant à des personnes décédées. Si cette situation est marginale à l’échelle nationale, elle concerne particulièrement certaines régions, la plus touchée d’entre elles étant la Corse.

La Corse est effectivement le territoire le plus marqué par cette situation de désordre. Le fameux arrêté d’André François Miot, droit spécifique historique fondé par cet administrateur des départements du Liamone et du Golo, reposait initialement non sur le principe de l’exonération, mais sur une absence de sanction en cas de non déclaration d’une succession fondée sur le double constat d’une indivision généralisée et d’une extrême pauvreté. La suppression, en 1949, de la contribution foncière sur laquelle reposait la liquidation des successions a engendré une exonération de fait. Ce désordre foncier est générateur d’insécurité juridique et produit des effets économiques néfastes. L’absence de titres de propriété empêche d’abord les citoyens de recourir aux dispositions de droit civil relatives à la propriété immobilière. Elle entrave également toute possibilité d’accès à l’emprunt. La détention de biens par de multiples héritiers censés détenir des droits indivis concurrents dilue les responsabilités et rend plus difficile l’entretien des biens concernés. Tous ces éléments participent au délabrement du patrimoine immobilier et alimentent d’abondants contentieux dans les familles. Cette situation est également lourde de conséquences pour les autorités publiques, l’État et les collectivités territoriales. Le recouvrement de l’impôt sur le foncier et surtout des droits de succession relève d’un parcours du combattant. du combattant. Ainsi, le montant des droits de succession collectés en Corse s’élevait à 6,7 millions d’euros en 2013, premier exercice ayant suivi la fin de l’exonération totale des droits, qui sont depuis lors recouvrés à hauteur de 50 %.

Il est important de rappeler que la loi de 2017 faisait suite à la volonté exprimée par le législateur à plusieurs reprises sur ce sujet. Celle de 2002 établissait des périodes transitoires, le temps que la situation foncière soit normalisée civilement.

Il ne devait pas perdurer au delà de 2027, mais ses statuts ont été modifiés et sa pérennité est désormais assurée, tant le travail de reconstitution des titres de propriété sera long. Il est logique que les mesures incitatives découlant de la loi du 6 mars 2017 soient prorogées au delà de 2027 pour que tous les moyens soient engagés afin de mettre un terme à cette situation préjudiciable.

L’objet de cette proposition de loi est tout simplement de proroger les mesures de la loi du 6 mars 2017 jusqu’au 31 décembre 2037, au lieu du 31 décembre 2027. Si le travail du Girtec a connu une progression fulgurante depuis la promulgation de la loi en 2017, on est encore loin d’atteindre l’objectif de normalisation ayant justifié la prorogation des mesures dérogatoires pour une période décennale. Alors pourquoi dix ans ?

J’espère emporter l’adhésion du plus grand nombre d’entre vous, mes chers collègues, mais aussi celle du Gouvernement, qui connaît bien cette problématique. Je finirai en m’adressant à vous, madame la secrétaire

faute de procédure associée. J’ai sollicité à plusieurs reprises la Chancellerie pour obtenir, sinon un décret d’application, du moins une circulaire pour permettre aux notaires de mobiliser cet article. En vain

J’ai été obligé de signer la vente de la moelle de mes os […] à un prix de détresse qui ne représente ni la valeur morale ni la valeur matérielle. J’ai emporté avec des larmes, en quittant le seuil, les vestiges de ma mère et les reliques de ma jeunesse. Le désordre foncier, particulièrement prégnant en zone rurale, n’est pas une fatalité. L’application du principe d’équité justifie que la représentation nationale s’empare à bras le corps de cette question et y réponde pleinement et justement.

En février 2017, ce même texte avait obtenu un soutien massif dans cet hémicycle, ainsi qu’à l’Assemblée nationale, où j’espère que le texte prospérera rapidement cette fois ci encore et tout

Toutes les conditions procédurales et politiques sont donc réunies pour parvenir à l’adoption de ce texte. Je vous demande d’en prendre acte et je compte sur votre soutien pour renouveler l’opération de 2017 en adoptant largement cette proposition de loi.

Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, il y a sept ans déjà, en 2017, notre assemblée adoptait la proposition de loi visant à favoriser l’assainissement cadastral et la résorption du désordre de propriété. Nous examinons aujourd’hui sa prorogation, sur l’initiative de notre collègue Jean Jacques Panunzi. Cette proposition de loi témoigne ainsi de l’intérêt et du travail continus des parlementaires pour répondre à une problématique ancienne, celle du désordre foncier et de l’irrégularité cadastrale en Corse. Depuis plus de deux siècles, la Corse se caractérise en effet par une situation foncière tout à fait spécifique, du fait de l’absence de titres de propriété, de l’inexactitude du cadastre ainsi que de la pérennisation de nombreuses situations d’indivision successorale dans des proportions bien plus importantes que sur le reste du territoire français. Cette situation est la conséquence de mesures dérogatoires en matière d’imposition des successions instaurées par l’arrêté Miot de juin 1801. Ce dernier, abolissant les sanctions pour défaut de déclaration de succession, a entraîné l’arrêt du règlement des successions pendant près de 200 ans sur le territoire corse.

dont les cinq premiers visaient à accélérer la résolution du désordre foncier en Corse. Nous avions, à l’époque, adopté ces cinq articles, dérogatoires du droit commun, en limitant leur application pour une durée de dix ans, c’est à dire, en l’état actuel du droit, jusqu’au 31 décembre 2027. Les articles 1 et 2 prévoyaient la sécurisation de la possession des biens par le recours à la prescription acquisitive ainsi que l’assouplissement des règles d’indivision afin de faciliter la résolution des situations d’indivision successorale. Pour mémoire, l’article l’article 1 facilitait le recours aux actes notariés de notoriété acquisitive pour attester de la possession d’un immeuble situé en Corse et abaissait à cinq ans le délai pour porter une action en revendication contre un tel acte. En complément, l’article 2 assouplissait les règles de majorité pour la gestion des indivisions constatées par un acte de notoriété acquisitive, en abaissant à la majorité simple, contre une majorité de deux tiers dans le droit commun, le seuil requis pour accomplir les actes d’administration indispensables à la bonne gestion du bien. La loi du 6 mars 2017 portait également trois mesures d’ordre fiscal, très importantes, visant à inciter à la résolution des successions et à la reconstitution des titres. L’article 3 a étendu pour dix ans une exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit, applicable sur l’ensemble du territoire national lors de la première mutation postérieure à la reconstitution des titres de propriétés y afférents. Outre la prorogation du dispositif, la loi du 6 mars 2017 a également rehaussé le niveau de l’exonération, la faisant passer de 30 % à 50 %. L’article 4 de cette même loi prorogeait par ailleurs le régime dérogatoire en matière de droits de succession, mis en place en 2002, qui applique aux biens immobiliers situés en Corse une exonération partielle des droits de succession à hauteur de 50 %. Enfin, l’article 5 rétablissait, toujours pour une durée de dix ans, une exonération des droits de partage de succession sur les immeubles situés en Corse, qui était précédemment applicable jusqu’en 2014. Cinq ans après l’entrée en vigueur de ces mesures, la commission des lois a considéré que leur bilan était encourageant. D’une part, ni le Conseil notarial de Corse ni le ministère de la justice n’ont observé de difficulté contentieuse du fait de l’application des mesures dérogatoires au droit civil créées par le texte. D’autre part, il est établi que la reconstitution de titres ainsi que la résolution des situations d’indivision ont progressé depuis l’adoption de la loi, au regard de la baisse du nombre et de la proportion de parcelles appartenant à des propriétaires décédés. Le groupement d’intérêt général pour la reconstitution des titres de propriété en Corse estime ainsi que 1 868 titres ont été créés depuis l’entrée en vigueur de la loi du 6 mars 2017, ce qui représenterait au moins 15 000 parcelles. Ces efforts de titrement ont permis de réduire de 4,6 points de pourcentage la proportion de parcelles appartenant à des propriétaires présumés décédés, celle ci s’établissant désormais à 30,4 %, ce qui est encore beaucoup trop.

Le coût de ces exonérations semble par ailleurs raisonnable, le montant de l’exonération régie par l’article 3 de la loi du 6 mars 2017 étant évalué à 20 millions d’euros. Toutefois, à date, la quantité et la difficulté des dossiers de reconstitution des titres n’ont malheureusement pas permis la régularisation du désordre foncier et successoral sur l’île.

C’est encore beaucoup trop, pour ne pas dire énorme, au regard de la statistique nationale, qui avoisine les 100 % de parcelles titrées. Cette situation à tout le moins singulière entraîne une grave insécurité juridique ainsi que d’importantes conséquences pour la puissance publique.

et conduit, trop souvent, à la dégradation des biens par défaut d’entretien ainsi qu’à la multiplication des contentieux intrafamiliaux. Nous sommes en Corse, chers collègues, et nous savons à peu près ce que cela signifie Pour la puissance publique, le désordre foncier se traduit par une perte de recettes fiscales, qui limite la capacité des collectivités à entretenir leur territoire. De plus, il convient de rappeler que l’absence de propriétaires identifiés constitue un risque en matière de bonne administration, mais aussi de sécurité civile, en raison de la dégradation et du manque d’entretien progressif de nombreuses parcelles rurales et montagneuses,

Pour toutes ces raisons, il semblerait aussi improductif que dangereux de se satisfaire de l’extinction des mesures créées en 2017 d’ici à trois ans. Devant le constat que l’achèvement des travaux de titrement nécessitera encore plusieurs années, la présente proposition de loi tend à proroger de dix ans les dispositifs visant à accompagner et à faciliter la résolution du désordre foncier et l’assainissement cadastral de la Corse.

la résolution des situations d’indivision persistantes, la protection du droit de propriété sur l’ensemble du territoire français ainsi que la régularité du cadastre, sont des objectifs atteignables si nous poursuivons les efforts engagés, dont les bénéfices dépassent le coût des exonérations temporaires induites par ce texte. En conséquence, la commission des lois a fait le choix d’adopter la proposition de loi de notre collègue Jean Jacques Panunzi en l’état et vous invite aujourd’hui à faire de même, considérant que l’adoption de ce texte permettra de poursuivre le travail vertueux engagé par tous les acteurs locaux depuis maintenant sept années. La parole est

depuis près de deux siècles, la Corse connaît une situation foncière dégradée du fait de l’absence de titres de propriété, de l’inexactitude du cadastre et d’un niveau d’indivision successorale considérablement plus important que sur le reste du territoire français. L’origine de cette situation remonte à l’arrêté du préfet Miot de juin 1801, qui encourageait les administrés à régulariser leur situation par la mise en place de mesures fiscales exceptionnelles. Il s’agissait en réalité de les dispenser de toute sanction en cas d’absence de déclaration de succession. Malheureusement, en supprimant ces sanctions, l’arrêté Miot a dissuadé les familles corses de déclarer leurs successions pendant près de deux siècles. deux siècles plus tard, la Corse se caractérise par une situation cadastrale et foncière particulièrement dégradée. Ainsi, plus de 300 000 parcelles sont détenues par des personnes physiques nées avant 1910, soit 30 % des parcelles de l’île. par une inexactitude cadastrale, qui entraîne l’existence de biens non délimités sur 6,4 % des parcelles corses, contre 0,4 % sur l’ensemble du territoire.

ou au crédit, tandis que la sortie des indivisions peut se révéler très coûteuse ; d’autre part, pour les autorités, dans la mesure où les personnes publiques ne peuvent recouvrer l’impôt de manière satisfaisante, le problème se posant surtout pour la taxe foncière,

Cet outil, dont l’efficacité est reconnue et appréciée en Corse, fait actuellement l’objet d’un travail de réflexion, sous l’autorité du garde des sceaux. Il s’agit de le renforcer et d’assurer sa pérennisation budgétaire.

visent à faciliter le recours aux actes de notoriété acquisitive et aux règles de sortie de l’indivision, notamment par des mesures fiscales incitatives à la résorption du désordre de propriété. Il est important, mesdames, messieurs les sénateurs, de souligner que la loi de 2017 est un outil utile, qui répond à un besoin réel en Corse. Vous le savez, le Gouvernement a engagé durant deux ans des discussions resserrées avec les élus corses, notamment dans le cadre d’un comité stratégique. Sans surprise, ce sujet a été abordé à de nombreuses reprises, singulièrement par le sénateur Jean Jacques Panunzi, dont je salue ici l’engagement et le souci de trouver des réponses pratiques et rapides aux préoccupations quotidiennes des Corses. En prolongeant de dix ans les dispositifs pertinents de la loi de 2017, le Parlement facilitera le travail de reconstitution des titres, qui, bien qu’inachevé, progresse.

Malheureusement, malgré cette amélioration, la proportion des parcelles corses disposant d’un titre foncier régulier, de l’ordre de 70 %, est encore trop peu élevée pour que l’on puisse considérer que la situation est satisfaisante, en particulier au regard du même taux à l’échelon national, supérieur à 99 %. Les notaires le constatent, le cadre civil posé par la loi et les exonérations fiscales ont créé une dynamique incitant enfin les particuliers à chercher à résoudre les problèmes d’indivision qui courent depuis plusieurs générations. Malgré le bilan encourageant de la loi, des marges de progression importantes demeurent et appellent, selon nous, une action résolue de prorogation de la loi jusqu’en 2037. N’oublions pas que, au delà de ses implications juridiques et administratives, le désordre foncier en Corse revêt une dimension politique importante et contribue, d’une certaine manière, à la spéculation immobilière en soustrayant un volume significatif de foncier. Force est toutefois de reconnaître que ce dispositif dérogatoire est particulièrement important et qu’il convient de le sécuriser. C’est la raison pour laquelle nous ne devons pas nous priver d’identifier toute amélioration technique. Dans l’intervalle, il est de notre responsabilité collective de nous donner les moyens de contribuer au maintien d’une politique volontariste de la Nation en faveur de nos compatriotes corses.

doivent normalement prendre fin le 31 décembre 2027. Ce texte concerne très majoritairement la situation cadastrale de biens immobiliers situés en Corse.

ce qui a eu pour effet non seulement d’exonérer ceux ci des droits de succession, mais également de créer de nombreuses indivisions, inconnues de l’administration du cadastre et, par suite, des services fiscaux.

Presque deux siècles plus tard, cette situation a été confirmée et même aggravée par un arrêt de la Cour de cassation du 2 janvier 1992. La Cour y considérait que, faute de base légale de calcul, les droits de succession ne pouvaient pas être recouvrés. Dès lors, en Corse, même quand les successions étaient déclarées, la mutation des biens n’était pas taxée.

leur situation. Était ainsi prévue une exonération de moitié des taxes pour les successions ouvertes entre le 1 janvier 2013 et le 31 décembre 2027,

être rémunéré. Dans ces conditions, la réticence des propriétaires dépourvus de titres à déclarer une succession susceptible de leur occasionner des frais trop importants Nous en déduirons que la prorogation de dix ans demandée aujourd’hui par cette proposition de loi apparaît justifiée ; pour ma part, je la voterai.

Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, la Corse se trouve dans un désordre cadastral et foncier très particulier. En 2016, il était estimé que 35 % des parcelles cadastrées y étaient enregistrées comme appartenant à des propriétaires décédés.

de 1801, dont le principe était l’absence de sanction en cas de défaut de déclaration de succession, porte une large part de responsabilité dans cette situation inextricable de désordre foncier.

d’une part, les propriétaires ne sont pas en mesure de jouir totalement de leurs droits ; d’autre part, les pouvoirs publics ne peuvent pas pleinement recouvrer l’impôt. Face à cette situation de profonde insécurité juridique, la loi du 6 mars 2017 est venue apporter une réponse concrète au désordre de la propriété en six articles, dont les cinq premiers se rapportent à la Corse ou à l’ensemble du territoire national. L’article 1 consacre le recours aux actes de notoriété acquisitive notariée ; l’article 2 assouplit les règles de majorité applicables en matière d’indivision. Les articles 3 à 5 comportent, quant à eux, des dispositions de nature fiscale. L’article 3 prévoit notamment une exonération de droits à hauteur de 50 % de la valeur de l’immeuble lors de la première mutation à titre gratuit d’un bien nouvellement titré ; l’article 4 proroge de dix ans l’exonération partielle de droits de succession applicable aux immeubles situés en Corse ; enfin, l’article 5 rétablit, jusqu’en 2027, l’exonération des droits de partage de succession sur les immeubles

du désordre de propriété pour le développement de la Corse, le groupe Les Indépendants est convaincu de la nécessité de poursuivre le mouvement vertueux de titrement du foncier ainsi engagé ; il votera donc à l’unanimité en faveur de cette proposition de loi.

parler des spécificités de la Corse n’est ni un vain mot ni un péché d’autocentrisme – la proposition de loi de notre collègue Jean Jacques Panunzi l’illustre à bien des égards.

Cela permit d’adapter la fiscalité nationale des successions à la situation corse, déjà marquée par la prédominance des indivisions et des successions orales.

et des dommages collatéraux qu’elle allait causer pendant plus de deux siècles, tant l’intérêt s’attachant à l’absence de déclarations favorisa le maintien des propriétés en indivision. Pendant plus de deux siècles donc, à cette spécificité législative s’ajouta la particularité de l’inaction : deux cents ans qu’aucune solution juridique satisfaisante soit envisagée pour résoudre l’un des principaux fléaux de l’île, qui a lourdement pesé sur son économie, dégradé le foncier et ruiné des villages entiers.

sans compter les abondants contentieux qu’elle alimente au sein des familles. Et cela reste un handicap très lourd à l’heure où nous cherchons à revitaliser un monde rural qui se désertifie, où tant d’habitations tombent en ruine alors que nombre de personnes, souvent jeunes, voudraient s’y installer et y vivre. Ce mal, conjugué aux problématiques de spéculation immobilière et de logement, nous oblige à rappeler le lien indéfectible des Corses à leur terre, mais aussi les tensions multiséculaires qu’il a fait naître

Face à tant d’incurie, face à une telle carence législative, il fallait trouver un remède pour résorber le désordre foncier, pour que ce mal générateur d’insécurité juridique cesse de nuire dramatiquement à notre territoire.

est précisément l’enjeu de la loi de 2017, qui a permis la mise en place de mesures dérogatoires et transitoires pour une période de dix ans, de manière à accélérer la reconstitution des titres de propriété en vue d’un retour, à terme, au droit commun. Sept ans après sa mise en œuvre, si les effets de cette loi laissent apparaître un bilan satisfaisant – 1 868 titres ont été créés, pour 15 000 parcelles – l’horizon d’achèvement des travaux de titrement semble encore lointain.

Si les mesures adoptées en 2017 et prolongées par ce texte permettent, sous réserve d’un accord politique, de résorber lentement et péniblement l’effet de siècles d’ingérence, elles ne sauraient se faire à droit constant.

Nous demandons donc à sortir d’un système dérogatoire, non sécurisé constitutionnellement et, par définition, transitoire, au profit d’une situation pérenne qui stabiliserait l’architecture au plan civil, par l’octroi de compétences adaptées. C’est précisément en raison du risque d’inconstitutionnalité qui pèse sur la résolution législative des problématiques spécifiques à notre île que l’inscription de la Corse dans la Constitution est nécessaire

la difficulté qu’auront les Corses à conserver leur patrimoine à la fin du régime transitoire, compte tenu de l’augmentation proportionnelle de l’impôt sur les successions, corollaire de l’augmentation des prix induite par la spéculation immobilière. Aussi, mes chers collègues, avec mes collègues du groupe Union Centriste, je vous propose d’adopter ces dispositions qui contribueront à la mise en ordre du foncier dans l’île, tout en gardant à l’esprit que la Corse mérite, comme dans bien d’autres domaines, le solutionnement à droit constant de la question foncière. La parole

cette proposition de loi sert essentiellement à prolonger des mesures dérogatoires, de nature fiscale et civile, afin de résoudre les difficultés liées au désordre de propriété qui touche la Corse.

bien au delà. Nous faisons depuis plusieurs années le constat d’une raréfaction et d’une complexification des ressources fiscales et financières des collectivités territoriales, faisant des finances locales un système imprévisible, illisible et inaccessible, notamment pour les élus des plus petites collectivités.

la non mise à jour du cadastre empêche le recouvrement d’impôts locaux, nos collectivités insulaires se retrouvent extrêmement pénalisées dans leur autonomie fiscale. Parlons d’autonomie, justement depuis le 27 mars dernier, avec le vote de l’Assemblée de Corse, nous sommes sur le chemin d’un projet de loi constitutionnelle portant statut d’autonomie pour la Corse. La résolution du problème du cadastre et du désordre de la propriété démontre, si besoin en était, la véritable nécessité d’un droit à la différenciation de nos territoires à la particularité, dirait notre collègue Paulu Santu Parigi. Nous constatons donc la pertinence du grand projet à venir pour l’autonomie de la Corse, qui permettra une adaptation à ses spécificités

Notre groupe, vous le savez, est toujours en faveur d’une simplification passant par une différenciation locale. Nous sommes tout autant des défenseurs de la construction des politiques publiques sur des faits et des évaluations. Avant de discuter

Si le besoin de résorption du désordre de propriété est un constat partagé, nous nous demandons si les moyens déjà mis en place ont fait l’objet d’une évaluation.

Mes chers collègues, nous saluons les avancées pour les citoyens et la sécurisation juridique de leurs biens, en particulier par la procédure de prescription acquisitive et la limitation des délais de recours. Je rappelle seulement que la prescription acquisitive établie par notaire requiert une possession continue, paisible et publique pendant trente ce sujet aurait pris toute sa légitimité en aval des discussions sur l’autonomie de la Corse. Nous sommes plus réservés sur l’opportunité de prolonger des mesures n’ayant pas fait l’objet de retours d’expérience. Nous voterons toutefois ce texte, qui répond à l’objectif de résorption du désordre cadastral, dans l’attente du débat sur le projet de loi constitutionnelle, lequel apportera des solutions structurelles en accordant à la Corse – nous en formons le vœu – le pouvoir d’adopter des lois adaptées

Le premier proroge, de 2027 à 2037, un dispositif facilitant le recours aux actes notariés de notoriété acquisitive sur le territoire corse le second proroge des exonérations fiscales incitant les particuliers à régler les questions successorales laissées en suspens depuis trop d’années. Parce qu’elle reconduit un régime dérogatoire et crée des situations exceptionnelles, d’un point de vue tant territorial que temporel, cette proposition de loi devrait avoir quelque chose d’insatisfaisant. Une lecture froide et trop stricte de ce texte nous laisserait même avec une forme de pessimisme. Pour autant, le droit n’est pas une chose froide et inerte, comme on le croit trop grossièrement ; nos lois sont toujours le fruit d’un contexte social et historique. Les quelques mois que j’ai déjà passés dans cet hémicycle n’ont cessé de me le rappeler. Légiférer n’est pas une science mécanique, mais un travail d’anticipation, parfois plus ou moins adroit, qu’il faut adapter et toujours corriger en fonction des circonstances et de leurs spécificités.

elle a conduit, au fil des années, à accumuler des situations d’indivision complexes, liées à l’absence de titres de propriété. Dès 2017, le Parlement a adopté des mesures visant à régler ces difficultés la loi du 6 mars 2017 a consacré dans le code civil les actes de notoriété acquisitive issus de la pratique notariale permettant de constater que la possession d’un bien répond aux conditions de la prescription acquisitive. Cette pratique a été ouverte pour dix ans, jusqu’en 2027. L’échéance se rapproche, et nous constatons qu’il reste beaucoup à faire. Notre rapporteur a dressé un état des lieux de la situation suffisamment explicite et convaincant. Nous souscrivons donc à la prorogation proposée, en espérant que ces dix années supplémentaires de recours aux actes notariés de notoriété acquisitive, ainsi qu’aux dispositifs fiscaux, permettront d’arriver au bout de ce processus.

la proposition de loi qui nous est présentée a pour objet de reporter de 2027 à 2037 le terme des dispositifs transitoires institués par la loi du 6 mars 2017 visant à favoriser l’assainissement cadastral et la résorption du désordre de la propriété.

devaient permettre de résoudre le désordre foncier qui y prévaut. Héritée d’un arrêté de 1801 abolissant les sanctions pour défaut de déclaration de succession, grève, aujourd’hui encore, la sécurité juridique des individus et entrave le développement des collectivités territoriales, qui ne peuvent recouvrer l’impôt de manière satisfaisante.

de la délégation sénatoriale aux outre mer, de coordonner la rédaction de trois rapports procédant à une évaluation inédite de la situation des droits fonciers dans l’ensemble des territoires ultramarins.

Elles résultent de dévolutions successorales non réglées, voire non ouvertes, sur plusieurs générations. À l’instar du groupement d’intérêt public pour la reconstitution des titres de propriété en Corse, le Girtec, des mécanismes novateurs ont été conçus pour venir à bout de ce problème majeur. Je pense aux agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des 50 pas géométriques. Ces outils de coopération entre l’État et les communes, d’un vaste chantier de régularisation des occupations foncières, ont vu leur durée de vie prolongée plusieurs fois par le Parlement. À Mayotte, la commission de l’urgence foncière, créée par le législateur en 2017, mais devenue opérationnelle en 2019, a pour objectif d’apporter une aide aux particuliers qui souhaitent s’engager dans une démarche de régularisation foncière en mettant en œuvre une procédure de titrement.

telles que l’exonération de 50 % des droits dus lors de la première mutation à titre gratuit d’un bien immobilier, concernent l’ensemble du territoire français. Le présent texte contribue à rappeler à notre assemblée qu’à droit constant il est absolument impossible de résoudre ce désordre foncier.

Pour des raisons socio historiques et géographiques, ces territoires se trouvaient dans une situation cadastrale et foncière très dégradée, liée à l’absence de titres de propriété. Au delà de ses implications juridiques et administratives, le désordre foncier en Corse revêt une dimension éminemment politique, enracinée dans son histoire et exacerbée par le régime dérogatoire instauré par l’arrêté Miot du 10 laissant place à un régime fiscal transitoire. Je tiens à remercier le rapporteur André Reichardt pour ses travaux éclairants sur ce sujet au demeurant très complexe.

garanti. La sortie des indivisions peut, de plus, se révéler très coûteuse. Sur l’ensemble de l’île, l’accumulation des successions non réglées entraîne la détérioration

à la reconstitution d’un titre de propriété, exonération partielle des droits de succession et exonération temporaire des droits de passage sur les actes de partage de succession, à hauteur de deux fois et demie la valeur du bien.

Enfin, nous savons bien qu’à deux reprises, en 2012 et en 2013, le Conseil constitutionnel a censuré des mesures d’exonération des droits de succession sur les immeubles situés en Corse, estimant que le maintien de ce régime fiscal dérogatoire méconnaissait le principe d’égalité devant la loi et les charges publiques. Si le Conseil

Au regard des progrès soulignés par le Girtec et devant l’ampleur du travail qui reste à accomplir, nous voterons ce texte.

Mes chers collègues, l’ordre du jour appelle l’examen des conclusions des commissions mixtes paritaires chargées d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l’organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, deux mois après l’examen de ces textes en séance publique, je suis heureux de vous retrouver pour la lecture des conclusions des commissions mixtes paritaires sur le projet de loi relatif à l’organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre aux défis de la relance de la filière nucléaire et sur le projet de loi organique qui lui est associé. Je souhaite tout d’abord saluer la qualité et la fluidité des échanges que j’ai eus avec le député Jean Luc Fugit,

maintenir notre sûreté nucléaire au niveau d’exigence le plus élevé possible en l’adaptant aux enjeux de notre décennie et des décennies à venir. Le projet de réforme qui nous a été soumis modernise notre système de sûreté nucléaire pour faire face au défi sans précédent la relance du nucléaire en France, défi auquel la gouvernance de la sûreté doit, elle aussi, s’adapter. Le projet initial présentait cependant des risques qui nous ont conduits à ajuster le texte présenté par le Gouvernement.

de sûreté. Une séparation insuffisante risquerait en effet de placer l’expertise sous l’influence de la décision ou, inversement, de placer la décision sous l’influence de l’expertise

Le texte que nous examinons aujourd’hui évite ces deux écueils. Il traduit la distinction entre expertise et décision de manière concrète dans l’organisation des instructions, en rétablissant la volonté sénatoriale de consacrer une distinction entre le personnel chargé de l’expertise et celui chargé de la décision pour un dossier donné. Il assure la confrontation des doutes indispensable à la sûreté nucléaire, en garantissant que, pour chaque instruction, l’expert est distinct du décideur tout en évitant de créer une muraille de Chine au sein de l’ASNR, en prévoyant bien que l’expert et le décideur interagissent

La crédibilité et l’acceptabilité de la relance du nucléaire reposent sur cette exigence de transparence. Je me réjouis de constater que le texte adopté en commission mixte

Le texte que nous examinons prévoit toutefois que l’ASNR pourra faire exception à cette règle générale, notamment au regard de la nature des dossiers concernés ou pour favoriser la participation du public.

Je me félicite du maintien de cette commission dans le texte final, moyennant une modification de son champ d’action. Enfin, le quatrième risque du texte initial était relatif à l’association du Parlement et de la société civile.

afin de garantir que la lettre du règlement sera bien conforme à l’intention du législateur. En définitive, ce texte illustre la capacité de nos assemblées à parvenir à un accord dans l’intérêt commun

pour le calendrier des projets nucléaires, sans nullement amoindrir pour autant nos exigences en matière de sûreté. Le texte a donc deux objets principaux, la création d’une autorité unique de sûreté nucléaire et de radioprotection et l’adaptation des règles de la commande publique aux projets nucléaires.

autorité. Toutefois, je vous le répète, le processus ne fait que commencer. Je me suis engagé, comme Christophe Béchu l’avait fait auprès de vous, à suivre de très près la mise en œuvre de la réforme et à nommer rapidement un préfigurateur qui nous permettra de reprendre le travail opérationnel de rapprochement. donc un compromis parlementaire, un texte issu des deux chambres, qui ont réussi à se mettre d’accord sur les enjeux majeurs de demain. Bien évidemment, j’espère que les parlementaires ici réunis voteront ce texte, qui est le fruit d’un consensus réfléchi et abouti entre députés et sénateurs. Nous passons

nous voici, à la fin d’un long processus parlementaire, amenés à entériner la fusion de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) et de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN). Comme je l’avais dit il y a quelques semaines, ce texte constitue, à notre sens, une victoire idéologique dans le débat crucial sur la souveraineté énergétique de la France. Le parc électronucléaire français, produit de notre génie national patiemment édifié pendant des décennies, représente notre meilleur atout pour notre compétitivité comme pour les obligations de la France en matière de transition écologique. Sans clairons ni trompettes, notre pays fut, dans une indifférence quasi générale, le premier à entamer et à terminer sa transition énergétique. Alors que l’Allemagne se vautre encore dans une production charbonnière criminelle que d’autres États – je songe à la Pologne – s’inquiètent de leur dépendance à des sources d’énergie fortement carbonées, les Français disposent d’une énergie propre, bon marché et sécurisée. Nous ne pouvons que nous féliciter que le Gouvernement, après des années d’errance dramatique, se soit rangé à l’avis des scientifiques comme de l’opinion. La relance de notre parc électronucléaire est notre passeport pour une croissance décarbonée et durable. À cet ou loi Nouveau Nucléaire, aussi insuffisante soit elle, constitue un premier pas dans la longue reconstruction de notre indépendance nationale. Pour autant, le présent projet de loi n’exonérera le Gouvernement ni de ses errements passés ni de son passif. vous avez emprunté durant le précédent quinquennat des directions contradictoires, voulant d’abord réduire notre parc de centrales nucléaires avant d’annoncer, pressé par les signaux de vos erreurs,

Ce texte a provoqué les inquiétudes légitimes de certains acteurs et spécialistes de la filière nucléaire. Le Parlement devra, particulièrement lors de l’examen des textes financiers à venir, rester vigilant sur l’existence de moyens réels pour que la nouvelle autorité sa mission en toute sérénité et en toute efficacité. La sécurité nucléaire ne repose pas sur des normes de papier, mais sur des moyens humains, des agents compétents et intégrés dans le processus industriel de construction et de suivi des installations nucléaires. Néanmoins, nous jugeons cette fusion bienvenue. Nombre de pays bénéficiant également d’une industrie nucléaire développée ont fait le choix d’un système de sécurité unitaire, ne compromettant

travaux d’une commission mixte paritaire conclusive. Voilà, nous y sommes ! La gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection est cruciale à bien des égards. Notre ambition est de relancer notre puissance nucléaire. Comme je le disais en première lecture, il faut désormais transformer l’essai. Grâce à des mesures concrètes et pragmatiques, ce texte est une première pierre, une première pierre, celle d’une souveraineté énergétique retrouvée pour la France. Le présent projet de loi, très attendu sur ce volet, même s’il a eu du mal à trouver son chemin législatif, n’est finalement que la traduction juridique d’une volonté très claire. Nous avons besoin de trouver les bons équilibres quand il est question de notre énergie et de notre production d’électricité. Un nucléaire régénéré ira de pair avec des énergies renouvelables, efficaces et développées de manière pragmatique, l’un ne pouvant fonctionner sans les autres. La France a besoin de tenir sur ses deux jambes en matière énergétique. Notre pays va devoir faire face à de nombreux défis. Décarboner notre production énergétique participe par définition Il faudra nous adapter aux conséquences du changement climatique, qui rend vulnérable notre nucléaire. Nous devons adapter notre parc vieillissant et garantir la sécurité de ses installations, existantes et nouvelles.

Nous ne pouvons consentir à laisser la gestion de notre approvisionnement énergétique à d’autres puissances, qui plus est lorsque ce sont des puissances ennemies. L’Union européenne ne peut plus se soustraire à son besoin de puissance. La souveraineté énergétique en fait partie, et elle passera par la relance du nucléaire. Dans ce cadre aussi, une gouvernance efficace de la sûreté nucléaire et de la radioprotection est une condition de la réussite de cette relance. Les enjeux sont immenses et je tiens à saluer le travail du Sénat, en particulier de notre excellente commission

Comme en première lecture, le groupe Les Indépendants reste attaché à une distinction entre l’expertise et la prise de décision. La solution retenue semble correspondre à cet objectif. Nous y resterons très attentifs.

Ils constituent la force du nucléaire et de sa relance. Il est de notre devoir de faire en sorte que la création de l’ASNR permette également la mise en place d’un cadre de travail qui leur correspond.

Je pense que la recherche et l’innovation trouveront là une structure intéressante pour apporter le progrès dont a besoin la filière. Enfin, je le répète aussi, même si ce n’est pas le sujet du texte, nous devons consacrer les moyens nécessaires à notre transition énergétique ; le nucléaire en fait pleinement partie.

aucun de nous ici n’a oublié l’introduction pour le moins maladroite de ce projet de fusion entre l’IRSN et l’ASN par le Gouvernement,

menaçait de déposséder le Sénat d’un débat pourtant déterminant pour nos territoires, au vu de la répartition des centrales nucléaires à travers le pays. De fait, beaucoup d’entre nous percevaient que cette réforme posait de nombreuses questions, qui ne pouvaient trouver de réponse satisfaisante dans les délais qui nous étaient impartis. Heureusement, le Gouvernement a entendu raison et temporisé, car réformer un sujet aussi sensible dans la précipitation aurait entraîné une prise de risque inconsidérée pour la sûreté nucléaire du pays. Ce temps, le Parlement l’a mis à profit pour se pencher plus en détail sur cette fusion potentielle, notamment grâce au rapport rendu en juillet 2023 par MM. Piednoir et Fugit pour le compte de l’Opecst, et aux travaux de nos collègues rapporteurs, MM. Martin et Chaize, dont je salue l’engagement en commission sur ce sujet. Ces travaux sont venus rappeler utilement les enjeux majeurs qui accompagnent la relance assumée du nucléaire pressurisés européens de type EPR2 ; évolutions technologiques telles que les SMR ; prolongation de la vie des réacteurs existants et augmentation de leur puissance ; gestion des déchets nucléaires adaptation des infrastructures au changement climatique et aux risques cyber ; enfin, démantèlement des centrales en fin de vie. Des difficultés inattendues peuvent par ailleurs survenir, telles que les problèmes de corrosion sous contrainte rencontrés en 2021 et 2022 sur certains de nos réacteurs. Par conséquent, les travaux à réaliser dans les prochaines années en matière de sûreté nucléaire sont voués à croître de manière importante, ce qui plaide à mon sens en faveur d’une seule entité issue d’un rapprochement entre l’IRSN et l’ASN. Je tiens néanmoins à rappeler que plusieurs conditions doivent être réunies pour la réussite de ce projet.

de garantir un niveau de transparence élevé pour que nos concitoyens continuent d’avoir confiance dans le nucléaire. Enfin, il faut procéder à des recrutements massifs

comme en témoigne le texte issu de la commission mixte paritaire, qui préserve les apports de notre Haute Assemblée tant sur la forme que sur le fond.

autorité et ses éventuelles modifications soient présentés aux parlementaires dans le cadre de l’Opecst. Ces acquis permettent de compléter une réforme ambitieuse

le chevalier au tablier de plomb, ainsi équipé contre toute radiation, a réussi à réveiller le nucléaire français, la Belle au bois dormant, longtemps assoupie à cause des mauvais sortilèges de la fée Carabosse, que certains ont parfois dépeinte sous les traits de Dominique Voynet. L’histoire pourrait s’arrêter là et la campagne, surtout normande, se retrouver peuplée de magnifiques châteaux de type EPR2, en attendant les SMR en vente dans tous les supermarchés. car il y a un « mais », quelques obstacles se dressaient encore sur la route du chevalier Nukleel. Ainsi, un mage fourbe avait imaginé un buisson touffu, capable de ralentir toute cavalcade trop rapide qui s’affranchirait du code de la route et des règles de sécurité. En imaginant deux structures différentes, réparties entre l’expertise et l’autorité, ce législateur des temps anciens voulait éviter toute précipitation au détriment de ladite sécurité. Et ce système, ce duo de sirènes d’alerte de l’IRSN et de l’ASN – vous noterez le souci de la rime – suscitait l’intérêt, pour ne pas dire l’envie, des royaumes voisins. Mais notre chevalier, héros de la geste nucléaire, n’a pas le temps de se faufiler dans le buisson, certes franchissable, mais à condition d’en respecter les codes. Il est en effet pressé par le danger, car l’empereur Photovoltaïque a déjà, à l’échelle mondiale, rapidement étendu son domaine

il a été décidé concernant les personnels chargés de l’une et de l’autre, que les uns ne seraient les autres que quand les autres ne pourraient plus être les uns, sans que les uns puissent pourtant jamais être les autres J’espère que vous avez suivi et, surtout, que l’ensemble des règles de fonctionnement de cette nouvelle entité sera consigné dans un livre magique,

Ce soir, mes chers collègues, nous actons de nouveau la rupture du dialogue, donc de toute possibilité de confiance, entre la société française et le monde du nucléaire. C’est la malédiction historique du nucléaire français.

ce projet de loi qui ne répond pas aux exigences de transparence démocratique, puisqu’il a été élaboré sur la base d’un rapport dont je rappelle que les conclusions ont été gardées secrètes.

réalité des faits –, vous avez fait le choix d’une procédure accélérée pour contraindre le travail législatif. Tout au long des débats s’est fait jour votre incapacité à démontrer les dysfonctionnements que vous imputez à notre système dual de contrôle de sûreté nucléaire. Vous n’avez fourni aucun document, aucune étude pour étayer la position du Gouvernement, qui prétend qu’un système unitaire serait plus performant. Même sur le plan économique, vous ne démontrez en rien l’opportunité d’un projet qui, dans un certain nombre de domaines, coûtera – vous le savez – bien plus cher C’est également un passage en force institutionnel, alors que toutes les instances consultées sur ce projet de fusion ont émis des réserves, voire exprimé une franche hostilité. Surtout, vous

SMR. Comment pouvez vous justifier la refonte intégrale d’un système qui a fait ses preuves, dans un moment aussi crucial ? Comment ne pas voir derrière cette fusion la volonté d’accélérer d’accélérer et de simplifier l’arrivée de nouveaux acteurs du nucléaire, alors que la sûreté des installations devrait être notre priorité absolue ? Comme de nombreux chercheurs l’ont indiqué, une proportion considérable des incidents graves résulte de causes organisationnelles, aussi bien à l’intérieur des entreprises et des agences concernées que dans les relations institutionnelles établies entre elles. Aussi, ce projet réalisé à la hâte, qui ne semble reposer que sur la volonté de bâillonner les experts et les chercheurs de l’IRSN, fait naître un risque pour l’ensemble de la population.

Cette phase ne doit se nourrir que de faits scientifiques et non de considérations économiques ou industrielles. Ce que vous proposez, je le redis, est Aujourd’hui, la production nucléaire est une activité hautement capitalistique. Les enjeux économiques liés aux décisions de démarrage ou d’arrêt des centrales sont donc prégnants. Si l’objectif de minimiser la durée de la phase de décision pour des raisons économiques peut parfois être compréhensible, nous considérons en revanche que l’impératif de sûreté doit toujours primer. Enfin, mes chers collègues, comment comptez vous renforcer la confiance de nos concitoyennes et concitoyens dans le programme électronucléaire, alors que ce texte conduira à une baisse drastique des impératifs de transparence des décisions, de droit à l’accès à l’information

passer en force un texte élaboré dans des conditions opaques par l’exécutif. Pour toutes ces raisons, nous voterons contre

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, la France s’engage dans une relance d’envergure, historique, de la filière de l’atome civil. À l’évidence, un tel virage ne se décrète pas sans préparer, adapter, ni renforcer les pièces maîtresses de la charpente qui porte l’édifice nucléaire de notre pays. La sûreté nucléaire est une d’entre elles. Reconnue dans le monde entier et forte de la confiance des Français, elle est peut être le pilier le plus solide de l’architecture actuelle.

J’entends qu’il faille adapter notre système de sûreté nucléaire à la forte progression de l’activité et au rythme soutenu des travaux qui s’engageront demain. Sans doute faut il raccourcir les circuits décisionnels et fluidifier les relations entre les acteurs ; sans doute faut il faire la chasse aux doublons ou aux dépenses inutiles – on en trouve toujours un peu partout chez nous. Mais faut il aller au delà, c’est à dire jusqu’à la fusion de l’Autorité de sûreté nucléaire avec l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ? Devons nous prendre le risque – c’est bien le mot qui convient

Au nom du groupe du RDSE, lors de la discussion générale en première lecture, j’ai exprimé les doutes que m’inspirait cette fusion menée tambour battant sur un sujet aussi sensible que celui de la sûreté nucléaire. L’enjeu est celui d’un risque potentiellement planétaire, rien de moins. Un hypothétique gain d’efficacité peut il justifier une prise de risque en la matière ?

J’estime notamment que faire d’un expert un décideur du jour au lendemain – et inversement – n’est pas un bon choix. Personnellement, je n’ai jamais rencontré un expert capable de décider. Les experts tirent leur force de leur acuité, de leur esprit d’analyse, de leur capacité à s’attacher aux détails.

La publication des avis d’experts en amont de la décision constitue le fondement de leur contre pouvoir, c’est à dire de leur capacité à influer sur la décision – n’en déplaise aux décideurs. Repousser la publication des rapports

faire de la France le premier grand pays industriel au monde à sortir de sa dépendance aux énergies fossiles. Il s’agit d’un défi d’une ampleur considérable. Pour le relever, nous devons nous appuyer sur la stratégie française pour

réduire nos émissions grâce à la production d’une énergie décarbonée ; baisser la facture pour les ménages ; tenir notre engagement à sortir des énergies fossiles participer à la réindustrialisation de la France – nos chantiers d’EPR2 seront les plus importants d’Europe ; enfin, renforcer la souveraineté énergétique de notre pays, dans un contexte géopolitique instable.

la relance du nucléaire va demander une montée en charge et en capacité inédite pour la filière depuis le plan Messmer. Il s’agit d’un changement complet

en précisant que cette distinction s’opère pour une instruction donnée et ne concerne que les dossiers pour lesquels l’instruction recourt à une expertise. Enfin, nous nous sommes accordés sur le projet de règlement intérieur de la future autorité, qui devra être présenté, comme les projets de modification, à l’Opecst.

dans les procédures de travail ; la mise en œuvre claire des dispositions sociales ; enfin, l’accompagnement du plan de recrutement massif, 100 000 postes devant être pourvus en dix ans – il s’agit, là encore, d’un défi colossal à relever. Pour toutes ces raisons, mon groupe se prononcera en faveur de ce texte de compromis. La parole

EPR. Quel dommage que, en 2015, le ministre de l’économie ait décidé de brader la branche énergie d’Alstom à l’américain General Electric, privant ainsi la France de ses turbines stratégiques

tenu des moyens de communication en réseau et du foisonnement de fausses informations, le meilleur moyen d’assurer la confiance est la transparence : plus l’organisation sera transparente, plus le doute sera éliminé. Dès lors, pourquoi faire l’inverse ? Pour faire plus vite,

et l’absence d’une évaluation sérieuse des risques d’une telle fusion ont conduit à retenir le statut d’autorité administrative indépendante pour le futur organisme, alors qu’une administration n’est pas un lieu approprié pour mener des projets de recherche. Cette question est tout particulièrement prégnante au vu de la part importante des moyens humains, mais surtout financiers, qu’il faudrait consacrer à la recherche au sein de la future autorité,

nuira à la viabilité de notre capacité de recherche, à la proportionnalité des mesures de sûreté, aux liens de sûreté et de sécurité entre

Pour réussir notre transition énergétique, nous aurons besoin de l’électricité nucléaire. Par cette réforme, nous allons retarder cette transition, désorganiser nos structures et nous exposer

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, les projets de loi ordinaire et organique que nous examinons comportent trois réformes techniques destinées à accompagner la relance de la filière nucléaire, qui a été actée par la loi dite Nouveau Nucléaire du 22 juin 2023. La commission des affaires économiques était chargée de l’examen au fond des articles 12 et 16 à 18 du projet de loi ordinaire, relatifs à la simplification des règles de la commande publique et au repositionnement du haut commissaire à l’énergie atomique. Elle s’est saisie pour avis des autres articles de ces projets de loi concernant la création de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. Je me félicite que la commission mixte paritaire soit parvenue à un accord. Ce ne fut pas facile, car la réforme était bien mal engagée. bien mal engagée. L’an passé, la commission des affaires économiques avait rejeté des amendements présentés à la hâte par le Gouvernement pour leur préférer une saisine de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques. C’était indispensable.

de la société Orano. Alors que le cycle du combustible nucléaire prend un tournant plus stratégique que jamais, il s’agit d’un progrès historique pour le contrôle parlementaire des décisions du Gouvernement comme des orientations de la filière nucléaire. concerne les articles 16 à 18, relatifs à la commande publique, je me félicite du maintien de deux facultés introduites par le Sénat pour les porteurs de projet : le critère de crédibilité des offres et le recours à des avenants. Ces souplesses additionnelles étaient demandées par la filière nucléaire. Nous sommes aussi parvenus à ajuster utilement le périmètre des souplesses administratives initiales

outre, nous avons obtenu de conserver l’obligation pour les porteurs de projet de notifier à l’État le recours aux dérogations aux règles de publicité et de mise en concurrence, dont le Gouvernement rendra compte à son tour au Parlement. Je suis convaincu que la simplification des normes doit s’accompagner d’un renforcement des contrôles. C’est une exigence économique pour prévenir toute dérive des délais et,, des coûts.

l’institution d’une commission de déontologie, ou encore le recours à un groupe permanent d’experts. Au total, les mesures que j’ai citées étant indispensables à la relance

demande du Gouvernement, l’examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique,

en matière de numérique, d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole. Ce projet de loi a fait l’objet d’une commission mixte paritaire conclusive le 4 avril dernier, ce dont le Gouvernement se réjouit. Cet accord est le fruit d’un dialogue constant et exigeant, notamment avec les rapporteurs Cyril Pellevat et Daniel Fargeot, dont je tiens à saluer le travail. Le droit français s’enrichit régulièrement des décisions prises conjointement avec les autres États membres. La création d’un cadre européen unifié est la meilleure protection et le meilleur moyen d’accompagnement que nous puissions garantir à nos entreprises et à nos concitoyens, et ce partout en Europe. C’est cette exigence de disposer d’un droit national conforme aux évolutions législatives européennes

Nous pouvons nous en réjouir et être collectivement fiers de ce bilan. Les Ddadue sont des objets particuliers et s’attellent bien souvent à des points très techniques. C’est la raison pour laquelle ce texte contient des habilitations à légiférer par ordonnance, dont je sais que les parlementaires ne sont généralement pas très friands. J’en conviens, mais soyez assurés, mesdames, messieurs les sénateurs, que le Gouvernement s’est efforcé de limiter au maximum leur nombre dans ce texte. De plus, nous avons veillé à ce que les délais octroyés soient raisonnables, tout en tenant compte de la complexité d’un certain nombre de dispositions à transposer.

d’utiliser les procédures de dérogation au principe du pays d’origine (PPO) afin que des règles protectrices des consommateurs français puissent s’imposer à des influenceurs installés dans un autre État membre de l’Union européenne, quand cela sera nécessaire et de manière proportionnée. Enfin, je me félicite que la commission mixte paritaire ait opté pour une durée d’habilitation de neuf mois. Ce délai est en effet nécessaire pour mener à bien les consultations juridiquement obligatoires, notamment celles de la Commission européenne et du Conseil d’État. Tout cela demande du temps et un tel délai nous permettra de mener à bien ces échanges.

Sur les plans économique et financier, je salue l’accord trouvé en commission mixte paritaire pour donner le temps nécessaire aux échanges entre la Commission européenne et les différentes parties prenantes. Plusieurs habilitations à légiférer par ordonnance sont données au Gouvernement, en matière tant de protection des consommateurs que de droit financier, pour protéger nos sociétés commerciales. Les amendements proposés par le Gouvernement aux articles 5 et 6 tendent à sécuriser, au regard de l’article 38 de la Constitution, les habilitations telles qu’elles ont été rédigées par la commission mixte paritaire. La première habilitation, à l’article 5, porte sur la directive relative à un meilleur équilibre entre les femmes et les hommes parmi les administrateurs des sociétés cotées, ou directive. La seconde habilitation, à l’article 6, permettra, quant à elle, d’adapter notre droit au règlement européen révisé sur les transferts de fonds, ou (TFR), qui renforcera considérablement notre dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux.

En matière de transition écologique, ce Ddadue traduit en droit français la définition de l’hydrogène renouvelable et de l’hydrogène bas carbone, éléments clés de notre politique de souveraineté énergétique. En matière de coopération judiciaire, je tiens à souligner l’importance du texte pour soutenir les dispositions renforçant notre lutte antiterroriste. Désormais, un égal accès des services répressifs de tout État membre aux informations disponibles dans d’autres États est garanti. En matière de protection sociale, plusieurs décisions de justice récentes portant sur le régime des congés payés avaient conduit le Gouvernement à présenter un amendement, sur lequel l’avis du Conseil d’État avait été demandé avant son dépôt, pour remédier à l’inconventionnalité d’un article du code du travail. Cette clarification est nécessaire pour tous les employeurs et tous les salariés. Enfin, en matière agricole, la gestion par les régions d’une partie des aides relevant du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) pour la programmation 2014 2022 est facilitée.

d’un cadre simplifié pour mener les actions de prévention des risques d’inondation prévues par la directive européenne du 23 octobre 2007. Des amendements ont été adoptés pour alléger et simplifier les procédures en la matière. mesdames, messieurs les sénateurs, nous pouvons nous féliciter que, sur ce Ddadue, les travaux menés de concert nous permettent de disposer d’un droit national conforme aux évolutions législatives européennes récentes, au service de nos entreprises et de nos concitoyens. Nous passons

à la place de l’établissement de l’élevage. À compter du 1 janvier 2026, les missions relatives à l’identification et à la traçabilité animale seront entièrement transférées aux chambres d’agriculture.

la prochaine mandature, issue des élections européennes du 9 juin prochain, sera déterminante dans un monde en plein mouvement, pour ne pas dire en pleine crise. L’Union européenne, ce n’est pas qu’un vœu ; ce sont des réalisations concrètes qui ont une influence sur la vie quotidienne de nos concitoyens, qu’il s’agisse de lutte contre le changement climatique, de guerre économique, ou de protection des citoyens.

De manière générale, ce texte, fortement teinté de dispositions sur le droit de la consommation et le droit des sociétés, sur les questions monétaires, financières et bancaires, traite de sujets marquants pour la vie économique. Il intègre également des avancées importantes, notamment l’incorporation dans notre droit du mécanisme d’ajustement carbone aux frontières, qui sont dans la droite ligne de la volonté exposée lors de la présidence française du Conseil de l’Union européenne. La bonne application de ces dispositifs, avec une période transitoire, permettra de donner corps aux impulsions que la France a pu donner au niveau européen. De même, les avancées concernant les systèmes d’échange de quotas d’émissions de l’Union européenne apportées par le Sénat sont préservées. Cela démontre, si cela était nécessaire, le sérieux du travail de notre commission spéciale. Par ailleurs, en première lecture, nous évoquions l’importance de l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Aussi, nous nous félicitons de l’élargissement de la liste des congés concernés Ce point a été conservé, ce qui va dans le bon sens. Enfin, j’aimerais évoquer deux nouveautés introduites par l’Assemblée nationale. Premièrement, l’article 33 met de l’huile dans les rouages de la distribution des fonds européens.

demandait plus d’ambition, au service des territoires. Cet article y contribue, mais nous devrons persévérer pour améliorer le système. La seconde nouveauté est l’article 35, qui permet de progresser dans les adaptations nécessaires de notre droit au sujet de la majorité numérique et de la lutte contre la haine en ligne. Nous devons rester intraitables et imposer nos propres règles : tout ce qui est interdit hors ligne doit l’être sujet particulièrement cher au groupe Les Indépendants. Nous le constatons, c’est à l’occasion de l’examen de ces textes, lors de leur intégration au droit interne, que nous pouvons, enfin, choisir l’Europe que nous voulons. C’est pourquoi le groupe Les Indépendants défend depuis sa création la fin de la surtransposition, qui est un mal bien français. Elle nous a pénalisés à de nombreuses reprises, notamment lors de la crise majeure qu’a récemment traversée le secteur de l’agriculture. La logique est la même pour les mauvaises transpositions ou les erreurs de transposition. À cet égard, je salue l’article 7 , qui, précisément, corrige des erreurs de transposition.

Je rappellerai que nos travaux préparatoires ont relevé des douze travaux d’Hercule : un seul mois entre la présentation du texte en Conseil des ministres et son examen initial au Sénat, sans étude d’impact exhaustive. Imposer à notre chambre de travailler dans la précipitation sur des sujets techniques qui méritent une analyse approfondie trahit un manque de considération extrême.

Je tiens à remercier le rapporteur pour l’Assemblée nationale, Ludovic Mendes, ainsi que Stéphane Vojetta, rapporteur pour avis, de nos échanges constructifs qui nous ont permis d’aboutir sur ces différents sujets. Je me réjouis du maintien de la totalité des apports sénatoriaux à

matière de droit agricole, j’ai maintenu à l’article 34 les clarifications concernant le rôle des chambres d’agriculture et de Chambres d’agriculture France en matière d’identification animale, agrémentées des améliorations proposées par l’Assemblée nationale. Je souhaite revenir sur un sujet particulièrement sensible de ce texte, celui de la réforme de la garde à vue, qui ne concerne rien de moins que le droit d’accès à un avocat dans la procédure pénale. Alors que le Gouvernement était alerté depuis plus de deux ans de la non conformité de nos règles de garde à vue au regard de la directive C de 2013, il a présenté au Parlement une réforme fort mal conçue et très approximative. En moins de quatre semaines, avec le président Buffet, nous avons œuvré pour faire en sorte que la clé de voûte de la procédure pénale ne s’effondre pas, en préservant la capacité de nos officiers de police judiciaire (OPJ) et de nos magistrats à mener sereinement leurs enquêtes. À ce titre, nous conservons la mention selon laquelle l’avocat choisi ou commis d’office doit se présenter sans retard indu. C’est là un aboutissement heureux pour le Sénat, qui a su rétablir la possibilité d’une audition immédiate. rapidement sur l’article 3, relatif à l’influence commerciale. Nous avons restreint le périmètre dans lequel le Gouvernement pourra agir par voie d’ordonnance, pour préserver l’essence même du texte voté à l’unanimité par nos deux chambres en juin dernier.

Le Gouvernement nous a donc proposé un amendement de compromis, concerté entre les deux chambres, qui reprend les apports du Sénat, notamment en renforçant les dispositions en la matière pour les entreprises d’État et autres groupements à caractère public.

Madame la secrétaire d’État, ne laisser que quatre jours au Sénat pour en étudier les termes relève d’une nouvelle avanie ! Aussi avons nous obtenu la suppression de l’article 3 autorisant le Gouvernement à légiférer par ordonnance

La déconnexion aurait été manifeste, alors que nous appelons tous de nos vœux la nécessaire simplification normative. J’ai donc défendu une réécriture plus en phase avec le fonctionnement quotidien de ceux qui produisent de la valeur.

qui peuvent être très importants : importants pour la cohérence de notre droit national avec le droit européen ; importants aussi parce qu’ils touchent souvent à des aspects concrets de la vie de nos concitoyens ou à la puissance de notre Union européenne. européenne. Je tiens une nouvelle fois à saluer le travail des rapporteurs de la commission spéciale et de la commission mixte paritaire. Si notre marge de manœuvre dans cet exercice de transposition est mince, le groupe écologiste du Sénat se félicite de voir quelques avancées inscrites dans le droit national.

Nous transcrivons avec ce texte une partie des mesures du pacte vert européen, le. Si quelques avancées ont pu être obtenues, c’est avec inquiétude que, plus généralement,

l’attitude du gouvernement français a été particulièrement critiquable. Obsédée par son nucléaire, la France a conclu des alliances néfastes avec les pays gaziers, réduisant de fait les objectifs européens en matière d’énergies renouvelables.

le Haut Conseil pour le climat constate qu’après plusieurs consultations et débats, ni la loi de programmation énergie et climat, ni la stratégie française énergie et climat, ni la troisième stratégie nationale bas carbone, ni le troisième plan national d’adaptation au changement climatique, ni la troisième programmation pluriannuelle de l’énergie n’ont été formellement adoptés, en dépit des obligations législatives.

Concernant l’interdiction des microplastiques, nous regrettons que la commission mixte paritaire ait maintenu l’inscription d’un moins disant environnemental dans le droit national, alors que nous proposions, comme d’autres groupes de notre assemblée, de supprimer cet article afin de conserver notre ambition en la matière.

les salariés n’accumuleront pas le même nombre de jours de congés payés selon la nature de leur arrêt maladie : accident du travail, maladie professionnelle ou arrêt simple. Il s’agit d’une mesure dangereuse, que nous dénonçons.

l’adaptation au droit européen prend du temps, mais ce temps est essentiel pour respecter le processus démocratique et pour tenter de rendre plus cohérent un texte qui porte sur des sujets particulièrement hétéroclites.

Ce texte contient d’autres aberrations en matière environnementale, comme les quotas gratuits des marchés de carbone. Cette supercherie purement financière a été créée pour contourner la TVA générée par les transactions sur les ventes de quotas carbone. C’est particulièrement vrai pour le secteur des transports, qui est justement le secteur concerné par la mise en place de ces quotas gratuits d’émission de gaz à effet de serre, et dont les émissions ont augmenté très fortement – 16 % en trente ans. Pour les autres secteurs, comme l’industrie, la réduction des émissions est largement due aux délocalisations, facilitées par une réglementation européenne qui fait supporter la production du CO2 par d’autres pays du monde avec des normes environnementales plus permissives.

Il nous est proposé une parité d’au moins 40 %, et ce sans sanction supplémentaire à l’encontre de ceux qui ne respecteraient pas cette obligation. Curieuse façon de traiter une grande cause nationale

Finalement, il apparaît qu’il est plus facile de porter atteinte au droit des prévenus que de porter le progrès social et écologique. Pour toutes ces raisons, même si nous reconnaissons

Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, le plus souvent examinés dans l’urgence, les projets de loi de transposition du droit européen ne recueillent pas, à mon sens, toute l’attention qu’ils méritent. Sous des abords relativement techniques, ces textes dissimulent des changements importants pour le quotidien de nos concitoyens, la vie de nos entreprises et de nos territoires. Le projet de loi dont nous débattons ce soir, et que l’on pourrait qualifier de fourre tout, contient même plusieurs je pense à la réforme de la procédure pénale. Ce volet est loin d’être anecdotique : il s’agit de revoir les conditions d’accès à un avocat lors de la garde à vue. Depuis deux ans, la Commission européenne alerte la France au sujet de ses manquements : je regrette que cette question fondamentale n’ait pu être débattue dans le cadre de l’examen d’un autre véhicule législatif – je pense notamment au projet de loi de programmation et d’orientation du ministère de la justice 2023 2027.

à un autre sujet, fruit lui aussi d’une construction transpartisane et consensuelle entre les deux chambres. L’article 3 habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour modifier notre loi du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale.

Le marché européen fermera progressivement la porte au moins disant environnemental. Une concurrence plus juste entre les entreprises européennes et celles des pays tiers pour une décarbonation de l’économie à grande échelle : voilà la bonne équation.

prouver l’inverse. Avec ce projet de loi de transposition, nous avons ce soir l’occasion de le dire clairement : oui, les normes européennes sont les bienvenues dans notre droit interne quand elles simplifient le quotidien de nos professions agricoles, lorsqu’elles rendent le droit du travail plus protecteur ou quand elles rétablissent un certain équilibre dans notre procédure pénale. Avant tout, je tiens à souligner le bien fondé de ce texte en matière de politique agricole, en insistant sur le Fonds européen agricole pour le développement rural.

Toujours est il que, lorsque les aides comprennent une contribution financière de l’État, les régions doivent obtenir au préalable la signature du représentant de l’État, ce qui allonge les délais de traitement. pour les décisions relatives aux financements apportés par l’État pour la programmation du Feader, donner la possibilité au préfet de déléguer sa signature au président du conseil régional et aux agents placés sous son autorité me semble une mesure bienvenue. Une telle tous. Les précisions relatives aux missions des établissements de l’élevage seront également utiles. Avec le présent texte, ces établissements peuvent se voir confier la délivrance et la gestion des matériels, des procédés et des documents d’identification et de circulation des animaux, ainsi que la collecte des données relatives à l’identification et à la traçabilité de ces derniers. Il s’agit là d’une transposition logique et pertinente, à la lumière du règlement européen relatif aux maladies animales transmissibles.

adopté en 2023 dans le cadre du Pacte vert. Enfin, ce texte de transposition rétablit un équilibre attendu par les avocats entre le respect des droits de la défense et la manifestation de la vérité pour l’efficacité de l’enquête.

paradoxal, la pratique judiciaire démontre que la présence de l’avocat en garde à vue renforce la valeur probante des propos recueillis. En résumé, ce texte assurera la mise en conformité de notre droit pour l’exécution des mandats d’arrêt européens

portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole. C’est bien sûr une bonne chose

: dans une Europe de vingt sept États membres aux histoires, aux géographies, aux économies et aux sociétés parfois très contrastées, l’harmonisation ne se fait pas toujours par le haut. Or le plus petit dénominateur commun européen n’est pas toujours la variable la plus appropriée à la France, en particulier en matière sociale et environnementale.

mixte paritaire. Échanges d’informations entre les polices, échanges numériques en matière pénale et de terrorisme, protection des libertés individuelles, application du Pacte vert avec le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières, la refonte du système d’échange des quotas d’émission, l’économie circulaire, les dispositions relatives aux la sécurité des produits de consommation vendus en ligne et la traçabilité animale : voilà autant de sujets sur lesquels nous pensons que l’Europe nous a fait avancer. Il en est de même pour la place des femmes dans les conseils d’administration et de surveillance. À cet égard, nous sommes rassurés qu’un accord ait pu,, être trouvé sur l’article 5. Avec ce projet de que l’Europe s’occupe de notre quotidien ; que l’Europe peut nous aider à relever les défis sociaux, environnementaux et économiques auxquels nous faisons face ; que l’Europe peut faire progresser les droits et libertés. L’Europe peut faire tout cela, à condition que la démocratie s’exerce pleinement en son sein. Les choix et les contraintes que

Sur ma proposition, nous avons mené un travail de coordination utile sur l’article 6, introduit à l’Assemblée nationale, qui détaille les obligations de déclaration de bénéficiaires effectifs de certains organismes. Enfin, à propos de l’article 6, qui suscitait le plus de difficultés, nous sommes parvenus à une position de compromis. La prolongation de six mois de l’habilitation à légiférer par ordonnance pour transposer le règlement Mica () sur les marchés de crypto actifs, introduite par le Gouvernement à l’Assemblée nationale, est maintenue dans ce texte. Le Gouvernement souhaitait

première lecture. En matière de transition écologique, je note que les apports sénatoriaux ont été conservés par nos collègues députés. À l’article 11, l’Assemblée nationale a ainsi préservé l’extension de l’obligation de contractualisation avec les éco organismes ou les systèmes individuels à l’ensemble de la chaîne de gestion des déchets de batteries : cette mesure n’est donc plus limitée aux seuls opérateurs de gestion de déchets. Aux articles 14 à 17, portant sur la refonte du système d’échange des quotas d’émission de l’Union européenne, les nombreux ajustements juridiques que nous avions opérés afin d’améliorer la qualité du projet de loi ont eux aussi été maintenus. Je pense par exemple à la meilleure prise en compte des incitations liées au prix du carbone lors de l’allocation de quotas gratuits au titre de l’utilisation de biocarburants par le secteur aérien. J’en viens à l’article 19, qui fait évoluer les modalités de calcul des émissions de gaz à effet de serre (GES), de l’hydrogène renouvelable et bas carbone,

Les modalités de calcul envisagées ne reprenaient pas l’ensemble du cadre européen prévu pour l’hydrogène. Or toutes les étapes liées à la production et à l’utilisation de cette énergie doivent être prises en compte.

lorsqu’un contrat de régulation économique est signé, l’Autorité de régulation des transports doit désormais apprécier le caractère modéré de l’évolution tarifaire, en moyenne, sur la durée couverte par le contrat. Je souhaite également saluer les apports de l’Assemblée nationale à cet article. Ils visent également à faciliter et à encourager la signature de contrats de régulation économique entre les concessionnaires et l’État. Je vous remercie